internationales. Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l'emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles

Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre

texte. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales

nous confirmons, par le dépôt de cet amendement, notre opposition au recours aux ordonnances ; nous sommes en cela cohérents. La préparation de ce projet de loi a été longue, puisque le processus a été engagé dès les Assises de la mobilité, qui se sont tenues à la fin de l'année 2017. Dès lors, nous ne comprenons pas

précisément, un certain nombre de ces mesures ont trait à des dispositions d'ordre social qui affectent le temps de travail, notamment, des jeunes marins. D'autres mesures touchent aux contraintes réglementaires en matière de protection de l'environnement, dont l'importance nous semble évidente. Nous estimons que les parlementaires doivent être saisis pleinement de ces sujets et nous demandons donc la suppression de cet article.

noté, madame la sénatrice, que vous êtes opposée par principe au recours aux ordonnances, dont je rappelle qu'il est tout de même prévu par notre Constitution. En l'occurrence, il s'agit très largement de mesures de transposition de textes internationaux

En effet, l'intérêt financier réel pour les armateurs de se passer d'un renouvellement de certification ne doit pas prévaloir sur l'intérêt général de la prévention des pollutions marines. Je tiens à rappeler la législation actuelle : le régime français prévoit que chaque navire doit faire l'objet, d'abord, d'une visite de mise en service, permettant notamment de délivrer les titres de navigation nécessaires à l'exploitation du navire, puis de visites périodiques. Pour des motifs de simplification et d'optimisation de l'emploi des ressources publiques, qui ne font- encore ! -que diminuer, et afin d'alléger les contraintes pesant sur les armateurs, le Gouvernement souhaite modifier ces dispositions pour mettre en place des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution sans durée de validité pour les navires d'une longueur de moins de 24 mètres, transport de passagers. Dès lors, les titres de sécurité, tout comme les certificats de prévention de la pollution, n'auront plus de durée de validité. Nous considérons à l'inverse que les certificats de prévention de la pollution doivent être régulièrement contrôlés et leur durée de validité limitée dans le temps. Une telle mesure paraît en outre antinomique avec l'étude d'impact, qui justifie la mesure par la nécessité de « recentrer l'action des inspecteurs de sécurité sur la réglementation liée à la protection de l'environnement ainsi que la protection des travailleurs, afin de répondre aux exigences internationales et communautaires

Il s'agit également de supprimer l'agrément spécifique des entreprises de travail maritime, qui fait aujourd'hui doublon avec l'inscription au registre des services privés de recrutement et de placement de gens de mer. Il s'agit enfin de garantir les conséquences d'une négligence des services de placement en cas de manquement à leurs obligations légales. Nous souhaitons, par cet amendement, préciser que l'armateur est responsable de l'ensemble des marins à bord, même s'ils par une société privée de recrutement, tant du point de vue du respect des temps de travail et de repos, ainsi que des conditions de travail, que pour le paiement des salaires et le rapatriement. Au sein de l'Union européenne, la recherche des coûts les plus bas a conduit certains États membres à développer des stratégies destinées

amendement, apporter une simple précision, dans la continuité de l'amendement précédent. Nous demandons que soit définie de manière plus précise la notion de « marin occasionnel », en fondant cette notion sur le nombre de journées passées en mer et donc par l'instauration d'un plafond. Cette notion est importante, car de cette qualification dépend l'application de régimes différents. Il importe donc que cette distinction soit à la fois opérante et la plus juste possible. Quel est l'avis de la commission ? Le juste possible. Quel est l'avis de la commission ? Le cadre de cette dérogation et ses conditions n'ont pas encore été arrêtés. Des concertations auront lieu entre le ministère des transports et les professionnels du secteur. J'ai eu l'occasion d'entendre les différents acteurs. Je trouve l'idée intéressante, mais

qu'il est nécessaire de s'assurer que ces conventions sont encadrées par un modèle de référence commun. Tel est le sens de cet amendement. Quel est l'avis de la commission ? Cette

monsieur le sénateur, que les conventions de stage sont encadrées par l'arrêté du 30 novembre 2017 fixant un modèle de convention de stage pour les élèves des lycées professionnels maritimes et des organismes agréés.

Guillaume Gontard. Par cet amendement, nous souhaitons garantir l'absence de lien entre les sociétés de contrôle privées et les armateurs, propriétaires ou exploitants du navire contrôlé. En effet, le présent article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnances le code des transports afin de soumettre à agrément les organismes de contrôle privés, dans le cadre de la délivrance des titres de navigation, et de préciser les tâches qui leur sont confiées. Si la procédure d'agrémentation peut effectivement être le gage de la qualité du respect de la réglementation, contrairement à la situation actuelle, nous comprenons bien,, la volonté du Gouvernement de déléguer encore un peu plus au privé, de cette manière, des missions régaliennes, lui permettant de faire des économies de court terme. Sans revenir sur l'opportunité de l'existence même d'organismes de contrôle privés, nous souhaitons simplement, par cet amendement, éviter les conflits d'intérêts et garantir l'impartialité de ces organismes privés dans leur mission, en imposant l'absence de lien entre l'organisme qui délivre des titres de navigation et les entreprises qui en bénéficient. Il s'agit donc d'un amendement de bon sens tendant à éviter toute collusion d'intérêts dans un domaine qui relève de la sécurité marine et, donc, de l'intérêt général. Quel

du trafic fluvial. Le foncier bord à voie d'eau doit donc être réservé, de façon prioritaire, aux usages fluviaux. Nous proposons donc que Voies navigables de France, ou VNF, puisse saisir de manière réactive les opportunités d'acquisition de terrains lui permettant l'accès à la voie d'eau pour sa mission de valorisation domaniale, ce qui permettrait de favoriser le développement de ce mode de transport. Cet amendement vise ainsi à préciser que l'un des outils juridiques permettant à cet établissement d'étendre ses possibilités d'acquisition de terrains est le droit de préemption.

à VNF, gestionnaire de la majeure partie du domaine public fluvial et navigable, chargé du développement des activités logistiques, industrielles et touristiques autour de la voie d'eau, de constituer des réserves foncières à ces fins et de mettre en cohérence les plateformes portuaires. Toutefois, le Gouvernement ne souhaite pas entraver l'action des collectivités locales qui disposent de ce droit. C'est pourquoi l'ordonnance prévue à l'alinéa 24 de l'article 37 modifiera les statuts de VNF afin de lui permettre de se voir déléguer ce droit par les collectivités. Votre amendement me paraît donc satisfait ; je vous propose donc de le retirer.

J'en viens à la question de la bonne utilisation de la voie fluviale sur le Rhône. Il s'agit d'un problème d'aménagement à quai dans le port de Fos, sur lequel des travaux sont prévus pour permettre l'accostage des barges fluviales.

Cette évolution à la hausse se justifie par l'apparition de la nouvelle réglementation applicable pour ce type de bateaux, l'ES-TRIN, qui impose des espaces et volumes additionnels tels que les zones de rassemblement et de circulation piétonne sur le pont, des sanitaires réduite, l'installation d'équipements de traitement des fumées de moteurs ou bien l'ajout d'un second groupe électrogène. Or la limite des 50 tonneaux de jauge au titre de l'exemption de permis d'armement ne permet pas de satisfaire les exigences de l'ES-TRIN sans diminuer très sensiblement la capacité du bateau de la rendre incompatible avec le trafic actuel des véhicules de nos passages d'eau, notamment aux heures de pointe. En conséquence, si cette limite à l'obligation de permis d'armement n'est pas adaptée aux contraintes actuelles, les départements et

de ces territoires et leur attractivité. Toutefois, en période estivale, on assiste à des phénomènes de concurrence déloyale entre, d'une part, des opérateurs assurant la continuité territoriale entre le continent et les îles tout au long de l'année, dans le cadre d'un contrat de service public, où la collectivité elle-même est en régie, et, d'autre part, des opérateurs saisonniers intervenant sur les mêmes trajets, mais de façon temporaire. Sans remettre en cause la légitimité de ces initiatives privées, il paraît nécessaire, comme solution de remplacement à la fixation d'obligations de service public prévues au code des transports, de prévoir la possibilité de mettre à la charge de ces entreprises privées une contribution à titre de participation

des établissements pour lesquels les villes peuvent lever une taxe de séjour la catégorie des ports de plaisance, puisque les riverains des côtes, en particulier les riverains des ports de plaisance, sont les premiers touchés par la pollution atmosphérique liée

par les riverains des ports n'est pas acceptable, c'est une certitude. La mesure que tend à insérer cet amendement revient à laisser à la collectivité le choix de proposer une augmentation de taxe de séjour afin de taxer indirectement les externalités négatives ou les effets négatifs produits par ces paquebots

est encombré- tant mieux pour les boutiques riveraines -de milliers de touristes occasionnels descendus de ces navires de croisière. La pollution est tout aussi réelle

ministre. On peut vouloir activer différents leviers fiscaux de taxes, mais je vous rappelle que, dans les ports, les navires de croisière payent déjà des droits de port, qui peuvent être modulés en fonction des normes d'émissions. Remarque intéressante ! Là, on ajoute des outils aux outils.

d'une seule travée. Mme la ministre nous dit que certains outils existent déjà. Profitons de la navette parlementaire pour améliorer la réflexion et montrons que le Sénat a envoyé ce signe positif, réaliste et pragmatique comme élément fort de la lutte contre le réchauffement climatique.

Je pense que cet amendement aurait été beaucoup plus pertinent si, au lieu d'augmenter les impôts, il avait eu pour objet de diminuer la taxe de séjour des bateaux ayant un mode

est ainsi libellé : La parole est à M. Éric Gold. L'objectif de l'amendement de notre collègue Jean-Pierre Corbisez est d'insérer un article additionnel prévoyant la mise au point d'une stratégie de transition énergétique dans le secteur maritime, avec un objectif de propulsion neutre en émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Il s'agit de mettre la loi en cohérence avec la décision prise au mois d'octobre dernier par l'Organisation maritime internationale, aux termes de laquelle, à compter du 1 janvier 2020, l'ensemble des navires commerciaux devront utiliser pour leur propulsion un fioul dont la teneur en soufre sera limitée à 0,5 %, contre 3,5 % aujourd'hui. Cette décision marque l'engagement de ce secteur dans un processus ambitieux de transition énergétique, dans un contexte d'explosion du trafic maritime depuis une vingtaine d'années. Rien que dans l'océan Indien, cette augmentation a été de a été de plus de 300 % depuis le début des années 2000. Il paraît donc indispensable d'anticiper cette situation en déclinant à l'échelon national et en concertation avec les acteurs concernés une stratégie nationale pour la transition énergétique des navires. Les trois

55 rectifié. En avril 2018, l'Organisation maritime internationale a pour la première fois adopté une stratégie de décarbonation ambitieuse, afin d'atteindre un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d'ici à 2030 et d'au moins 50 % à l'horizon 2050. Le projet de loi d'orientation des mobilités se donne pour objectif d'encourager le développement de la mobilité propre,

extrêmement vite. D'après certaines projections, surtout si des efforts sont consentis dans d'autres secteurs, cela pourrait représenter jusqu'à 20 % des émissions de gaz à effet de serre dans quelques décennies. Autant dire qu'il s'agit d'un sujet crucial et qu'il faut une stratégie.

concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % à l'horizon 2050 et de 40 % à l'horizon 2030. À ce stade, et dans l'attente d'un outil tel qu'un marché du carbone, qui enverrait des signaux économiques, nous plaidons en effet pour une réduction des vitesses,

devra formellement prévoir que VNF favorise et développe la concertation sur ses actions d'aménagement du territoire, avec l'État évidemment, mais aussi avec les acteurs économiques, au niveau régional, interrégional, national, voire européen. La concertation est la condition de l'efficacité économique de la voie d'eau. Cet amendement vaut pour le réseau national actuel. L'élu des Hauts-de-France que je suis anticipe en disant qu'il vaudra, rapidement

Cette précision est superflue et satisfaite. La rédaction du 1° de votre amendement ferait par ailleurs perdre son sens à la troisième phrase de l'alinéa 4 de l'article 37. Qui plus est, dans le cadre du canal Seine-Nord Europe, VNF ira bien entendu à la rencontre des acteurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur général de l'établissement et un certain nombre de responsables,

? Monsieur le sénateur, je vous confirme que les textes régissant VNF prévoient déjà une large concertation dans le cadre de son conseil d'administration, qui comprend des élus nationaux et locaux, ainsi que des personnalités qualifiées dans les domaines de la navigation intérieure, des transports, de l'énergie hydraulique, de la protection des milieux aquatiques et de l'aménagement du territoire. Il s'agit des articles L. 4312-1 et R. 4312-1 du code des transports. La concertation peut aussi se dérouler dans le cadre de ses commissions territoriales en régions, lesquelles comprennent des élus locaux et des acteurs publics et privés concernés par le domaine fluvial. Ce sont les articles D. 4312-19 et D. 4312-22 du code précité. De plus, les deux élus membres du conseil d'administration sont choisis parmi les élus locaux présidant des commissions territoriales des voies navigables. Au-delà du conseil d'administration, l'action de VNF se déploie naturellement sur le terrain, en accompagnement des territoires et des acteurs économiques.

au-delà des textes formels, il faut que VNF travaille avec les élus. Si quelqu'un ici connaît la liste des candidats à l'attribution d'une place de bateau en région parisienne, qu'il vienne me le dire ! Personne ne l'a jamais vue, les

dans le Pas-de-Calais a été assez exceptionnel, car il a été réalisé par la voie d'eau, avec l'accord du directeur territorial. Nous le constatons régulièrement et, sur un certain nombre de sujets, je peux témoigner du fait que VNF est plutôt facilitateur que bloquant.

cadre du grand projet structurant qu'est le canal Seine-Nord Europe. Je dois dire que nous avons travaillé en bonne intelligence, en bonne complémentarité. Le département avait mis à disposition de VNF ses agents chargés notamment d'un remembrement

vote. J'ai une proximité géographique avec le président Marseille. Il est vrai que nos deux départements ont souvent été, à travers les voies navigables, des territoires servants de la capitale, ce qui a posé un certain nombre de difficultés.

personne ne répondant aux appels d'offres ? Pour notre part, nous considérons que l'intérêt public doit être remis au coeur de la réponse politique. Comment répondre aux besoins croissants de mobilité, y compris dans des zones très denses ? Selon nous,

qu'une multiplication des opérateurs, cette option étant porteuse de risques lourds en termes de cohérence de l'offre et de sécurité. Pour toutes ces raisons, nous attendons du Gouvernement qu'il porte une autre voix auprès des instances européennes et qu'il fasse valoir l'exception française, pour les services publics et l'intérêt général. Nous souhaitons que ces secteurs soient soustraits au tout-marché et à l'exigence de rentabilité, incompatibles avec toute idée d'aménagement du territoire et, surtout, de solidarité. madame la ministre, mes chers collègues, nous abordons avec cet article 38 l'un des points durs selon nous de ce texte, comme vient de le souligner ma collègue Éliane Assassi. Vous le savez, nous sommes opposés à l'ouverture à la concurrence imposée par le règlement convaincus qu'elle va entraîner une dégradation de la qualité du service. Très souvent, ce sont en effet les entreprises moins-disantes qui remportent les appels d'offres. Certes, la concurrence des lignes de métro, de bus et de RER a été actée en Île-de-France, à différentes échéances, que je ne rappellerai pas ici. L'article 38 vise à permettre à la RATP de s'insérer parfaitement dans ce champ concurrentiel. Pour cela, vous modifiez les articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, qui définissaient jusqu'à présent les missions de la RATP. Il s'agit de lui permettre de créer des filiales en Île-de-France pouvoir exploiter de futures lignes et fournir d'autres services de transport- covoiturage, autopartage, vélos ou scooters en libre-service, billetterie, retrait de colis, etc. Bref, on élargit son périmètre pour une rentabilité tous azimuts, si j'ose m'exprimer ainsi. Pour l'heure,

Pour nous, cette filialisation de la RATP, au détriment d'une entreprise unifiée, est une véritable attaque contre le service public. Les salariés de la RATP, avec qui nous discutons, savent très bien que l'ouverture à la concurrence n'est qu'un prétexte pour imposer une productivité accrue, laquelle se traduirait par des centaines de suppressions d'emplois, la remise en cause des conditions de travail, un recul des droits, et ce au nom de la compétitivité. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de l'examen de l'article 39. Pour l'heure, vous l'avez bien compris, nous sommes fondamentalement contre cet article.

38. Nous abordons ici la question de l'avenir de la RATP dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Pour faire face à ce changement d'organisation des transports urbains en Île-de-France,

Ainsi, l'ensemble de l'offre va faire l'objet d'une stratégie d'allotissement par Île-de-France Mobilités, ce qui mettra brutalement fin au monopole de la RATP pour l'exploitation des lignes de bus. De l'aveu même des représentants de cette entreprise, ce changement sera extrêmement brutal. Nous y reviendrons lors de l'examen d'autres articles. Sur le fond, nous estimons que le morcellement de l'entreprise historique, qui sera obligée de recourir à la filialisation de ses activités du fait de la politique des autorités organisatrices

sur le nouveau pacte ferroviaire -, de définir l'offre de transports publics. Moi, je considère que c'est aux collectivités de définir les offres de service public, et donc aux autorités organisatrices. Nous avons donc effectivement une différence d'approche.

n'avons rien préparé, rien mis en place, ce sera désastreux pour le personnel, comme pour l'entreprise de transports publics. La parole est à Mme Laurence Cohen,

sociale, qui a clairement permis d'éviter des dégâts trop importants sur le statut des agents. Il y avait en effet une vraie volonté, comme on le voit ici, de casse de certains statuts et de précarisation des travailleurs. Cette perspective de filialisation

s'effectuera. Après de nombreuses réunions de concertation avec les représentants des salariés de la RATP et du secteur en général, nous vous proposons un cadre social de haut niveau pour accompagner cette ouverture à la concurrence. Ne nous trompons pas de débat

qu'il lance pour l'exploitation des lignes la clause dite de la « société dédiée ». En effet, l'instauration de telles clauses empêcherait de fait l'EPIC RATP, en tant que tel, d'exploiter ces lignes, organisant ainsi son démantèlement progressif et, à terme, L'entreprise historique serait ainsi obligée, pour pouvoir répondre et poursuivre l'exploitation d'un service qu'elle opérait déjà avant, de filialiser cette activité, participant ainsi à son éclatement. Nous considérons que cette pratique de « société dédiée », qui tend à se généraliser, n'apporte aucune plus-value en termes de qualité de l'offre. Le législateur doit donc encadrer son utilisation pour qu'elle ne soit pas utilisée comme un outil de déstabilisation de l'opérateur historique. Pour toutes ces raisons, nous proposons d'interdire ces pratiques qui nous apparaissent discriminatoires. Quel

sous la forme juridique qui lui paraît la plus adaptée aux lignes de services de transport qu'elle doit mettre en concurrence. Par ailleurs, la commission a validé la possibilité pour la RATP de constituer des filiales sans condition de forme juridique particulière, ce qui offre de la souplesse à l'ensemble des acteurs, notamment à la RATP. La commission émet un avis défavorable madame la ministre, en France, de définir le cadre juridique adapté pour s'assurer de l'équité de la concurrence et obtenir le maximum de transparence, ce que permet notamment une filiale. L'avis est donc défavorable.

nous proposons que la capacité de filialisation, accrue par cet article concernant la RATP, soit corrélée à la forme juridique de la filiale. Nous rejoignons là des débats que nous connaissons bien dans cet hémicycle, l'examen du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire sur le maintien ou non de capitaux à 100 % publics au sein des opérateurs historiques. À nos yeux, la forme de l'EPIC est la plus sécurisante, car elle est intrinsèquement liée à l'exclusivité de capitaux publics, l'évolution de capital ne pouvant passer que par le changement de statut, et donc par la loi. Afin de sécuriser la création de filiales et d'encadrer leur activité, nous proposons donc de limiter cette possibilité à la création de filiales sous la forme d'EPIC, évitant ainsi la dilution de l'opérateur historique dans une myriade de sociétés à capitaux publics et privés qui capteraient des décennies d'investissements publics financés par l'impôt de nos concitoyens depuis des années. Le contexte du projet de loi Pacte, récemment discuté au

parole est à M. Guillaume Gontard. Nous souhaitons que les filiales créées par la RATP pour répondre aux appels d'offres dans le cadre de la concurrence ne puissent exercer statutairement que des activités en lien direct avec leurs différentes missions, et non en lien indirect, comme le prévoit le présent article.

parfois même en se faisant concurrence, construire, aménager des réseaux, exploiter des lignes et fournir d'autres services de transport. Jusque-là, nous sommes à peu près d'accord ... Mais elle peut également exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ces différentes missions, notamment toute opération d'aménagement et de développement connexe aux infrastructures de transport. Nous considérons pour notre part qu'il n'appartient pas à la RATP, ni même à ses filiales, de devenir aménageur. Être opérateur de transport, c'est déjà une mission lourde, avec des besoins et des enjeux suffisamment pressants pour ne pas s'écarter de ses missions d'intérêt général. Cette course à la diversification, dans des secteurs où la RATP n'a pas de compétences propres, nous paraît particulièrement hasardeuse.

pour les services réguliers de transport routier, le 31 décembre 2029 pour les services réguliers de transport par tramway et le 31 décembre 2039 pour les autres services réguliers de transports guidés. Enfin, pour les Enfin, pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes, le monopole se termine à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024. Nous souhaitons en finir avec toute injonction de libéralisation qui pénalise les usagers et les territoires. à M. Mathieu Darnaud. Les conditions d'ouverture à la concurrence pour les réseaux routiers d'Île-de-France envisagées comportent de nombreux risques. Une solution d'ouverture progressive, équitable et efficace doit être trouvée, en concertation avec l'ensemble des transporteurs. Progressive, une solution optimisée et gérable pratiquement semblant possible sur une période allant de 2022 à 2026. Équitable, car il faut qu'une ouverture progressive intervienne avec, pour chaque vague, un équilibre entre les opérateurs. Opérationnelle, les transferts de contrats entre opérateurs nécessitant la mise en oeuvre de dispositifs afin de permettre le transfert de salariés entre entreprises ayant des cadres sociaux distincts. Ces dispositifs devront être déclinés par des accords sociaux devant être adoptés avant le transfert des contrats. qu'il faut définir les vagues en tenant compte à la fois des ouvertures des nouvelles lignes de métro, des réorganisations nécessaires des réseaux permettant de passer d'une logique d'opérateur à une logique de bassin de vie et des événements internationaux qui seront organisés par la France, en particulier les jeux Olympiques de 2024. Cet amendement vise donc à assurer les meilleures conditions d'ouverture à la concurrence des réseaux routiers franciliens. L'amendement

de prévoir une certaine progressivité et, surtout, des modalités de suivi pour veiller à un juste encadrement du processus. Dans cette perspective, l'amendement a pour objet de reporter la date de la première ouverture à la concurrence

le nouveau système à mettre en place en effectuant des expérimentations afin de pouvoir en analyser les retours, y compris en ce qui concerne l'encadrement social des salariés. Ce n'est que sous le bénéfice de telles expérimentations qu'une ouverture globale de ces marchés pourra se faire dans le cadre d'une concurrence socialement régulée et économiquement non faussée. Les

ailleurs, aucune demande n'a été formulée par Île-de-France Mobilités pour repousser l'ouverture à la concurrence. L'AOM se prépare, et cela commencera dès 2022 avec le réseau Optile.

Les autres amendements ont pour objet de revoir les calendriers d'ouverture à la concurrence, que ce soit pour mieux aligner les calendriers d'Optile sur ceux de la RATP ou pour lisser l'ouverture dans le temps. Je comprends cette préoccupation. J'ai eu l'occasion d'échanger sur ce sujet à plusieurs reprises avec la présidente d'Île-de-France Mobilités,

est l'avis de la commission ? L'article 8 de la loi relative au Grand Paris prévoit que des élus des collectivités territoriales siègent au conseil de la Société du Grand Paris.

est à Mme la ministre. L'objet de cet amendement est de prévoir un avis conforme de l'Arafer sur la rémunération de l'activité de gestionnaire d'infrastructure.

de l'Arafer. Quel est l'avis de la commission ? La commission se félicite que ce sujet important puisse être traité dès l'examen du projet de loi au Sénat. Nous avons travaillé en collaboration avec le Gouvernement sur ce sujet et j'ai échangé à de nombreuses reprises avec les différentes parties prenantes.

va, selon moi, renforcer le déséquilibre régional entre les départements en matière d'investissement dans les infrastructures de transport. Je sais que telle n'est pas votre analyse, madame la ministre.

particuliers et entreprises, qui continuent à financer la Société du Grand Paris, au travers notamment de la taxe sur les surfaces de bureaux et de la taxe spéciale d'équipement. Si le calcul du montant de la taxe sur les surfaces de bureau, étendue aux parkings commerciaux, intègre des modulations selon les territoires en fonction de critères économiques et sociaux, ainsi que selon la proximité ou l'éloignement de la zone dense, le montant de la taxe spéciale d'équipement Il est totalement anormal qu'un habitant de grande couronne, qui passe en moyenne deux fois plus de temps dans les transports qu'un habitant de la zone dite dense et subit chaque jour le cauchemar des incidents récurrents sur les lignes du RER, s'acquitte du même montant

Compte tenu de la situation financière de la Société du Grand Paris et des besoins de financement du Grand Paris Express, une telle évolution n'est pas souhaitable à court terme. Le débat pourrait avoir lieu lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, après que certaines questions d'importance auront été tranchées en concertation avec l'ensemble des acteurs. Je pense en particulier à la

profitera à l'ensemble des habitants de la grande couronne, notamment en renforçant les liaisons de banlieue à banlieue, en désaturant des lignes de RER existantes et en favorisant les relations de pôle à pôle entre la petite et la grande couronne. S'agissant du financement de la Société du Grand Paris, je pense qu'il ne faut pas fragiliser son modèle économique. J'entends la nécessité de différencier la contribution des territoires,

la construction et l'aménagement des sites de maintenance et de remisage de modes de transport- bus, tramway, tram-train, métropolitain. Il s'agit, selon ses promoteurs, d'aller vite pour préparer l'ouverture à la concurrence. Nous ne partageons pas cette volonté d'aller vers un recours généralisé aux contrats globaux. nous laissent par ailleurs assez dubitatifs. D'un côté, pour l'exploitation du service public, l'allotissement et la multiplication des acteurs seraient le gage de la performance. De l'autre, pour la construction des sites de maintenance, le principe de l'allotissement serait insupportable, car synonyme de rigorisme administratif et de perte de temps. Nous voyons donc bien que chacun voit midi à sa porte, et que les arguments se retournent en fonction des intérêts du moment. Pour ce qui nous concerne, nous considérons que les principes des marchés publics doivent être respectés et que la concurrence est incompatible avec les principes du service public. Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement est contraire à la position de la commission. Nous souhaitons que cette dérogation au principe de l'allotissement prévue à l'article 38

du Gouvernement ? Il me semble que cette mesure spécifique à Île-de-France Mobilités n'a pas nécessairement vocation à être codifiée dans le code de la commande publique et aurait pu rester dans la partie non codifiée de la loi d'orientation des mobilités. Toutefois, je m'en remets à la sagesse du Sénat.